Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, je souhaite que nous saluions la mémoire du président du Parlement européen, David Sassoli, qui est décédé hier. personnifiait, par ses qualités propres et dans l'exercice de ses responsabilités, les valeurs de l'Union européenne. C'était un homme de libertés en tant que journaliste, il connaissait plus que tout autre le prix de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Il était libre d'esprit, indépendant, peu enclin à suivre les mots d'ordre, d'où qu'ils émanent. C'était un homme intrinsèquement attaché au parlementarisme : il n'aura eu de cesse, pendant la pandémie de covid- et nous avions échangé sur ce sujet -, d'éviter que la démocratie ne soit mise entre parenthèses, de rappeler sans relâche les prérogatives du Parlement européen et d'appeler à la responsabilité de chacun, pour que l'urgence ne justifie jamais que l'on outrepasse ou que l'on traite avec désinvolture la représentation parlementaire. Comme président du Parlement européen, il fut un homme à l'écoute de l'ensemble des sensibilités politiques représentées, y compris les plus éloignées de la sienne. En témoignent les nombreux hommages à la suite de sa disparition, en provenance de tous les États membres et de tous les bords politiques. C'était un Européen de convictions. Issu de la vieille Europe, passionnément italien, c'est-à-dire pétri d'une histoire européenne, il a incarné ce qui nous unit, la démocratie, l'État de droit, les droits de la personne, mais aussi cette culture en partage, à la fois si évidente et si difficile

C'était un homme courageux qui a tenu à exercer ses responsabilités jusqu'au bout, malgré la maladie. Sa détermination suffit à forcer l'admiration. Alors que nous entamons la présidence française du Conseil de l'Union européenne, dans son volet parlementaire, par la réunion à partir de demain au Sénat de la Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires (Cosac), j'ai souhaité que le Sénat lui rende hommage.

Chacun sera attentif au respect des uns et des autres et à celui du temps de parole. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour le groupe Union Centriste.

est exposée à un autre risque : une pandémie démocratique ou présidentielle. Nul ne saurait s'en satisfaire Notre pays a pris des mesures pour les élections municipales et, avec le recul de cette expérience, pour les élections départementales et régionales. Quelles sont les mesures prises pour l'élection centrale, l'élection présidentielle, afin de faciliter les opérations électorales et de permettre une véritable campagne À l'instant présent, mes chers collègues, il n'y en a pas, et un comité de pilotage, aussi sympathique ou qualitatif qu'il soit, ne saurait en tenir lieu. En l'état de la circulation du virus, une vraie campagne, nous le percevons tous, passera par l'audiovisuel, par les chaînes de télévision, par les débats et très peu, objectivement, par des meetings ou la distribution de propagande. Nous ne pouvons pas traiter ce sujet par la voie d'amendements sur le projet de loi relatif au passe vaccinal que nous sommes en train d'examiner, puisque, vous le savez tous, l'élection présidentielle obéit à des dispositions organiques. Ma question est donc la suivante : allez-vous, madame la ministre déléguée, mesdames, messieurs les membres du Gouvernement, déposer un projet de loi organique, dans quel délai et avec quel contenu, pour éviter une pandémie de la démocratie ?

possible, en permettant la pleine expression des candidats mais aussi l'accès le plus direct de chaque citoyen à la campagne électorale. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, ont souhaité la mise en place d'une instance de dialogue et de liaison, qui mette autour de la table l'ensemble des services de l'État, les partis politiques les candidats déclarés à l'élection présidentielle. Ainsi, les questions relatives aux incidences de la pandémie sur l'organisation de l'élection présidentielle pourront être traitées de façon collective, dans un esprit de responsabilité partagée. Les travaux dudit comité de liaison seront pilotés par une personnalité indépendante, M. Jean-Denis Combrexelle. Cette commission aura vocation à traiter les aspects strictement sanitaires touchant à l'élection présidentielle. Ce comité de liaison élaborera, dans ce cadre, un vade-mecum, un protocole spécifique aux réunions politiques, comme cela avait déjà été fait en 2021. Il abordera aussi la question des protocoles sanitaires dans les bureaux de vote. Je conclurai en remerciant toutes les personnes qui font vivre la démocratie en tenant les bureaux de vote lors des élections. Si le ministère de l'intérieur organise les élections, c'est grâce à ces personnes, et notamment aux élus et aux bénévoles que celles-ci peuvent se tenir. Je les salue ! veiller à » sans nous indiquer de délai, alors qu'il y a une urgence : ce n'est pas convenable ! Dans ces conditions, notre groupe proposera aux autres groupes du Sénat de se concerter sur une proposition de loi organique afin de traiter, notamment, les questions de la double procuration, du dédoublement des bureaux de vote lorsque ceux-ci sont trop chargés, et surtout des obligations spécifiques à prévoir pour ouvrir un espace suffisant de débat dans les médias télévisuels.

L'école est un lieu sensible. L'école maternelle, en particulier, est un lieu d'apprentissage de la socialisation, ce qui rend impossible, physiquement, l'isolement des élèves ou le respect de tous les gestes barrières. L'école peut donc être aussi un lieu de propagation de la pandémie. Ce que nous ne savions pas il y a dix-huit mois, nous le connaissons mieux aujourd'hui, au moment où nous vivons la cinquième vague de cette pandémie. Dès l'instant que vous avez fait le choix, de maintenir ouvertes les écoles, comment ne pas comprendre le vaste mouvement social unitaire qui se prépare pour demain ? Les revendications des enseignants et de tous ceux qui environnent l'école sont justifiées, et les associations de parents d'élèves les soutiennent. Comment ne pas comprendre ce message, au moment où la situation devient intenable dans nos écoles, dans les familles et dans nos collectivités ? Ce dont il est question aujourd'hui, si nous conservons l'école ouverte, c'est mettre en perspective une nouvelle approche du sujet pour les deux ou trois années à venir. Cela devrait appeler le gel immédiat des suppressions de postes d'enseignants, ce qui ne semble pas être le cas au regard des cartes scolaires qui se préparent. Cela devrait appeler des recrutements nouveaux, pour assurer les remplacements dans les classes. Cela devrait appeler une ambition nouvelle pour le développement de la médecine scolaire. Cela devrait appeler, enfin, une politique de soutien à des investissements nouveaux avec les collectivités, pour installer, par exemple, des purificateurs d'air dans les classes. Pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, les suites que vous entendez donner à ces revendications ?

que les réponses soient à la hauteur des enjeux. L'école à des besoins nouveaux. Sachons relever ensemble ce défi

depuis deux ans, nous vivons avec la covid-19. Alors que la majorité des Français a fait preuve d'une grande responsabilité dans la lutte contre la propagation du virus, la radicalisation d'une minorité est incontestable. Nous constatons avec gravité que près de 1 200 maires, parlementaires et autres élus ont été pris pour cible en 2021. Malheureusement, le début de l'année 2022 n'est pas en reste. Dernier exemple en date l'agression dimanche dernier du député de Saint-Pierre-et-Miquelon, Stéphane Claireaux, devant son domicile, par des manifestants opposés au passe vaccinal. Les intimidations, les menaces, les actes de violence doivent être condamnés et combattus avec force, au risque d'être banalisés. Ces comportements intolérables ne concernent pas nos seuls élus. Les soignants et les professionnels engagés jour et nuit pour sauver des vies en font aussi les frais : lettres de menace ; centres de vaccination tagués et vandalisés, quand ils ne sont pas criblés de balles comme à Nyons, dans la Drôme

Vendredi dernier, c'est le responsable du centre de vaccination de Munster, dans le Haut-Rhin, qui a été agressé à la sortie de son établissement. Madame la ministre, la montée de la violence à laquelle nous assistons doit être fermement combattue.

s'engager pour les autres, quelle que soit l'instance concernée et quel que soit le mandat. Je veux saluer cet engagement, qui est au coeur de la démocratie, au coeur de la citoyenneté. Je veux d'ailleurs rappeler ici que la grande majorité des élus locaux sont bénévoles. sont bénévoles. En ma qualité de ministre chargée de la citoyenneté, je ne peux qu'être sensible à l'alerte que vous lancez, et que nous sommes nombreux à soutenir, sur l'augmentation substantielle des agressions qui ciblent les élus. Selon les chiffres du ministère de l'intérieur, au cours des onze premiers mois de l'année 2021, les violences contre les élus ont augmenté de 47 % et les outrages de 30 %. Ce sont 162 parlementaires et 605 maires ou adjoints qui ont été victimes d'atteinte volontaire à l'intégrité physique. Je connais l'engagement sincère et puissant de la Chambre haute à l'égard de nos élus, et le Gouvernement, bien évidemment, le partage. Derrière ces chiffres, il y a des réalités et des vies, des vies qui font vivre la démocratie. Défendre l'intégrité des élus est fondamental : le débat, oui la controverse, oui ; la violence et la menace, jamais ! Monsieur le sénateur, vous avez aussi mis en avant la situation des soignants, qui depuis 2019 luttent avec acharnement contre la pandémie mondiale. Je ne peux que vous rejoindre : il est honteux de voir nos soignants, qui sont mobilisés, agressés ! En Guadeloupe, département dont vous êtes l'élu,

qui découle de la multiplication de protocoles visant à gérer la crise sanitaire. Ce qui pose problème, c'est certes la propagation du virus mais aussi le caractère tardif de vos instructions et de vos revirements. La conséquence en est qu'une grève, qui s'annonce particulièrement suivie, aura lieu demain. Pouvez-vous nous dire quelle est la genèse de cette situation chaotique, à laquelle les élèves, les parents, les enseignants et les élus locaux sont confrontés ? Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les réponses à ces inquiétudes légitimes et à ce mécontentement réel, lesquels vont s'exprimer demain pour dénoncer l'inadéquation de protocoles qui épuisent les enseignants comme les familles ? Pouvez-vous nous dire, enfin, ce que vous comptez faire pour restaurer la sérénité dans ce climat particulièrement anxiogène et préjudiciable pour les enfants comme pour les enseignants ? La parole

monsieur le sénateur, pour votre question, qui me donne l'occasion de revenir sur la gestion de la crise sanitaire, en général, et sur la situation en milieu scolaire, en particulier, laquelle doit évidemment mobiliser toute notre attention.

! Nous avons dû aussi, et c'est la source des difficultés que nous avons, adapter notre politique de dépistage,

Monsieur le Premier ministre, je vous remercie de m'avoir fait l'honneur de répondre à ma question ! C'est toujours avec beaucoup d'intérêt et de respect que je vous écoute, même lorsque vous me tournez le dos

ou pour la gestion de la diffusion du virus l'immunité collective ? Le jour où vous aurez répondu à cette question, peut-être serez-vous davantage écoutés et compris par les parlementaires et par les Français

Depuis des semaines, le prix de l'énergie et des carburants augmente : +41 % pour le gaz ; +21 % pour les carburants ; +3 % pour l'électricité. Ces hausses ont conduit, à la fin de 2021, à un surcroît de dépenses mensuelles en énergie de 30 euros en moyenne par ménage par rapport à la fin de 2019. Les habitants des zones rurales et hyper-rurales sont particulièrement concernés par ces dépenses au regard des particularités géographiques et climatiques de nos territoires. Au coeur du Massif central, les hivers sont rudes, et les besoins en chauffage bien souvent plus importants qu'ailleurs. En Lozère, en Margeride ou dans les Cévennes, le véhicule personnel est indispensable au quotidien, que ce soit pour accompagner les enfants à la crèche ou à l'école, pour se rendre au travail, à un entretien d'embauche ou chez un médecin. Une fois de plus, ces augmentations sont vécues par nos concitoyens comme une double peine, car elles s'ajoutent à la perte de services publics de proximité et à l'absence de solutions de mobilité au quotidien. Oui, monsieur le ministre, les habitants de Balsièges, de Bédouès-Cocurès, de Saint-Pierre-le-Vieux ou de Pourcharesses doivent prendre leur véhicule pour acheter leur pain. C'est la réalité de nos territoires, le quotidien des Français Français ! Pour faire face à l'inflation, le Premier ministre a annoncé une prime exceptionnelle de 100 euros et la baisse de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Cependant, vous conviendrez que ces dispositifs ne permettront pas de compenser la hausse des tarifs sur l'année- notamment pour l'électricité, qui pourrait augmenter de 40 % au 1 février prochain.

? Quelles mesures spécifiques impulserez-vous pour la ruralité ? Notre République doit être présente aux côtés de tous ses citoyens, y compris ceux des territoires ruraux. La

Le Gouvernement a réagi en prenant un certain nombre de dispositions. La première vise les ménages les plus défavorisés. Le Premier ministre avait annoncé il y a quelques semaines-cela a évidemment été réalisé depuis -le versement d'un chèque énergie supplémentaire de 100 euros à 5,8 millions de ménages. Nous avons aussi mis en place une indemnité inflation, avec la volonté d'aider tous les Français gagnant moins de 2 000 euros net par mois, qu'ils soient ou non conducteurs de véhicule, pour les aider à faire face à l'augmentation des prix, et non seulement à celle des prix du carburant.

pour plafonner l'augmentation du prix de l'électricité à 4 % depuis le mois d'octobre 2021, et l'augmentation du prix du gaz au même montant que celui d'octobre 2021. Ces dispositifs sont actifs. Ils ont été validés par le Conseil constitutionnel et le Gouvernement les utilise pour limiter l'augmentation du prix de l'énergie. Ils ont un coût, pouvant représenter plusieurs milliards d'euros par an. nous les mettons en oeuvre parce que nous connaissons la situation que vous avez décrite. Je suis moi-même élu en Ardèche et ardéchois de naissance. Je sais combien l'usage d'un véhicule à deux ou à quatre roues est essentiel pour le quotidien, et combien il est nécessaire d'accompagner les ménages les plus fragiles face à cette flambée des prix de l'énergie.

Territoires. Monsieur le ministre, parlons cannabis ! Après des années de flou, le Gouvernement précise enfin la réglementation autour du CBD (cannabidiol), en interdisant par arrêté la vente de fleurs et de feuilles brutes de chanvre contenant ce CBD, la molécule non psychotrope du cannabis. Cette politique prohibitive, dont la faillite est évidente, pousse les milliers de personnes qui trouvent dans la fleur de chanvre un substitut au cannabis à se tourner vers les dealers au risque de leur santé : cela prouve, une nouvelle fois, que le combat pour la santé des consommateurs n'a jamais été votre objectif. Vous faites un vrai cadeau aux trafiquants Alors que tant de nos concitoyens trouvent dans ce produit de vraies vertus apaisantes et relaxantes, dans une société toujours plus sous tension, où la consommation d'anxiolytiques frise des records, vous les renvoyez dans l'illégalité. Vous freinez le développement d'une filière du chanvre prometteuse, répondant aux attentes sociétales et environnementales, permettant de développer tout le potentiel extraordinaire de cette plante complexe et pleine d'atouts. Nos agriculteurs ne vous remercient pas. En faisant prospérer la philosophie de l'interdit, celle-là même qui a perdu devant nombre de juridictions, de la Cour de justice de l'Union européenne à la Cour de cassation, et qui perdra peut-être demain devant le Conseil d'État, vous mettez en évidence l'étroitesse de la vision que vous avez du sujet, prisonniers de votre de votre politique de répression inefficace et dangereuse contre le cannabis. Nous sommes les leaders européens du chanvre, et nous allons prendre un retard considérable sur tous nos voisins européens, notamment sur les Allemands, dont le pragmatisme tranche avec votre dogmatisme paternaliste et contre-productif. Si la loi française interdit toute drogue à l'exception de certaines comme le tabac ou l'alcool, rappelons que le CBD n'est ni un stupéfiant ni un produit nocif pour la santé. Alors, monsieur le ministre, allez-vous revenir sur ces décrets ubuesques interdisant le CBD, comme l'ont fait la grande majorité de nos voisins européens ? La

Emmanuel Macron s'était présenté sous le costume d'un libéral moderne. En fait c'est un jeune conservateur, un type « Fillon II

La consommation d'anxiolytiques, qui a explosé avec la crise sanitaire, concerne plus d'un Français sur quatre. Voilà sans doute un vrai sujet de santé publique, qui mérite l'attention.

le feuilleton juridique français continue. Pendant ce temps, nos voisins européens accélèrent. Nous serons bientôt inondés de produits issus de pays où l'on ne devise pas sur les feuilles et sur les fleurs, comme nous seuls en avons le grand art.

maintient un haut niveau de protection des consommateurs et préserve notre politique ambitieuse de lutte contre les trafics de stupéfiants, comme l'a très bien expliqué M. Véran, il permet

Cet arrêté est donc une chance pour la filière, qui est aujourd'hui la première en Europe et qui dispose de grands donneurs d'ordre intéressés par ses produits, par exemple dans la cosmétique ou dans l'agroalimentaire. Ce marché représente 700 millions d'euros et 15 000 emplois. L'interdiction que vous mentionnez ne porte que sur les fleurs et les feuilles, qui ne peuvent être récoltées, importées et utilisées que pour une production industrielle. Elle est justifiée et je ne reviendrai pas sur les arguments développés par le ministre de la santé. Le CBD est un produit psychoactif.

à ceux qui nous suivraient, car c'est une question de responsabilité. Vous connaissez les outils qui sont à disposition. Nous sommes en train d'en discuter avec la Commission de régulation de l'énergie,

l'équation à cette crise énergétique n'a que des solutions perdantes, à l'heure actuelle, au regard de ce que vous venez de dire. La faute est en fait triple. C'est une faute économique, parce que cela va présenter un coût pour les finances publiques de l'ordre de 15 milliards d'euros.

appliqué le 3, modifié le 6, encadré par les préfets le 8 et assoupli le 10 par le Premier ministre, donne l'impression, selon les propos d'une directrice d'école, d'un mauvais jeu de société, dont les règles changent tous les deux jours. On avance lundi, on recule mercredi et, surtout, on n'y comprend plus rien ! Alors, ma question est très simple, monsieur le ministre : pourquoi tant d'impréparation ?

Ne vous inquiétez pas, cela ne m'empêchera pas de vous répondre si vous me laissez parler ! D'abord, il y a eu un conseil de défense le lundi qui a précédé la rentrée. Le lendemain, mardi, j'ai indiqué que les écoles seraient ouvertes le lundi suivant et que le principal changement concernerait le fait qu'il y aurait un ou plusieurs tests en plus de celui déjà existant. Les grandes lignes étaient donc

Tout cela est précis, complexe, doit être cohérent et a été travaillé par les hautes autorités. Dans la journée du 1 janvier, nous avons transposé ces mesures pour en faire le protocole. Le ministre de la santé s'est ensuite exprimé pour donner la doctrine en population générale, puis moi-même, sur l'école. Voilà le déroulé des

recul des savoirs fondamentaux, du « lire, écrire, compter » ; sortie de route du nouveau baccalauréat, devenu un maquis dans lequel se perdent les élèves ; absurdité du calendrier du contrôle continu, qui soumet les lycéens au stress de l'examen perpétuel ; effondrement de l'enseignement des mathématiques au lycée, dont vous projetiez pourtant le redressement ; circulaires caporalisantes sous lesquelles croulent les établissements, alors qu'il y a cinq ans vous annonciez leur autonomie ; jeunes professeurs toujours aussi mal payés, mal formés, toujours aussi peu considérés et malmenés par un véritable bizutage institutionnel ; démissions en masse et moral au plus bas ! L'attractivité du métier n'a jamais été aussi faible. Ils vont vous le dire demain avec force et avec le soutien des parents

finalement apparaître le « blanquerisme » pour ce qu'il est : un autoritarisme esseulé, expliquant largement « l'étrange défaite » dans laquelle sombre ce quinquennat en matière d'éducation La parole est à Mme Sylvie Robert, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. et Républicain. Ma question s'adressait à la ministre de la culture et de la communication. Annulations de spectacles, reports de dates, arrêts des tournées : telle est la situation difficile du spectacle vivant en ce début d'année.

Une relance soutenue était espérée en septembre 2021 ; malheureusement, cette reprise, marquée par un retour plus que timide du public, fut compliquée. La fermeture totale des lieux de culture pendant plusieurs mois n'y est peut-être pas pour rien ! Par-delà la déception ressentie par tous les acteurs culturels-nous la partageons -, il y a une réelle inquiétude pour l'avenir. Certes, les aides du Gouvernement et leur prolongation permettront au secteur de continuer à résister. Souhaitons-le, en tout cas ! Mais, monsieur le secrétaire d'État, ces lieux ne doivent plus être stigmatisés. Ils ne sont pas des espaces de contamination et les professionnels ont toujours été au rendez-vous, responsables : ils ont proposé et mis en oeuvre des protocoles sanitaires renforcés. Une véritable concertation entre tous les acteurs est attendue. Faisons-leur confiance et donnons-leur enfin la visibilité qu'ils réclament ! Nombre d'artistes et de techniciens sont en grande difficulté aujourd'hui, certains n'ayant pas retrouvé les plateaux depuis plusieurs mois. mois. Dans ce contexte difficile, l'année blanche des intermittents s'est arrêtée le 31 décembre dernier. Ma question est simple : avez-vous effectué une évaluation, et allez-vous prolonger le soutien jusqu'à l'été prochain ? La parole

Cette crise a très fortement affecté le secteur culturel partout dans le monde. Pour lutter contre le virus, il a fallu et il faut encore, à certains égards, limiter les rassemblements, alors que c'est le rôle et la force de la culture de rassembler, d'unir les Français et, par-delà la France, d'unir dans le monde entier.

Nos évaluations montrent que la grande majorité des intermittents a pu reconstituer leurs droits à la fin de l'année 2021, mais je vous le dis : tous auront un filet de sécurité durant l'année 2022. Nous réactivons les dispositifs sectoriels. Vous le voyez, madame la sénatrice : nous tenons à ce que la culture garde sa juste place au coeur de l'âme de notre pays.

La parole est à Mme Isabelle Raimond-Pavero, pour le groupe Les Républicains.

Daech a laissé derrière lui des combattants endoctrinés, des enfants et des adolescents ayant suivi tant des entraînements militaires intensifs qu'une formation aux codes et au discours de l'État islamique. Ces enfants ont grandi. Selon les services de renseignement, ils représentent une menace réelle et pourraient constituer une nouvelle génération de Plusieurs d'entre eux font l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées. Le milieu carcéral constitue également une menace et un défi majeur en matière de radicalisation, de prosélytisme passage à l'acte. Depuis le 26 juillet 2018, 1 976 individus inscrits au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste sont sortis de prison, dont 290 terroristes islamistes. Aujourd'hui, 1 073 individus en suivi actif sont incarcérés ; 71 d'entre eux d'entre eux vont sortir de prison d'ici à la fin de l'année, dont 13 individus condamnés pour terrorisme et 58 radicalisés, sans compter les libérations inopinées pouvant intervenir à tout moment. Plusieurs années ont passé depuis la défaite militaire de Daech en Irak et en Syrie. L'évolution de la situation de ceux qu'on appelle les « lionceaux du califat » et les sorties de prison des personnes radicalisées

pour gérer et anticiper tant ces situations concernant les « lionceaux du califat », restés sur place ou revenus en France, que les sorties de prison, qui font peser sur notre pays un risque terroriste élevé

Centriste. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, en tant que président du groupe interparlementaire d'amitié France-Asie centrale, je souhaite interroger le ministre des affaires étrangères à propos de la situation au Kazakhstan. La forte hausse du prix du carburant a donné lieu, au début de l'année, à un mouvement de contestation sociale de grande ampleur, qui s'est transformé en violentes émeutes, marquées par des échanges de tirs, le saccage de bâtiments publics et des pillages. Ces événements ont conduit le président Tokaïev à demander le soutien militaire de l'Organisation du traité de sécurité collective, afin de contrer ce que les autorités kazakhes ont qualifié d'« attaque terroriste ». Dans ce cadre, 2 000 hommes, essentiellement russes, ont été déployés dans le pays.

Ne faut-il pas se préoccuper de la présence de militaires russes dans ce pays, qui vient de célébrer le trentième anniversaire de son indépendance ? Quelles sont la position et l'action de la France et de l'Union européenne sur ce sujet ?

de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Nous souhaitons que toute la lumière soit faite sur les circonstances ayant conduit à ces événements tragiques. Par ailleurs, nous sommes attentifs au respect durable de la souveraineté et de l'autonomie d'action des autorités kazakhes, qui ont fait appel, vous l'avez souligné, à l'assistance de l'Organisation du traité de sécurité collective. Un contingent, en grande majorité russe, a donc été déployé dans le pays pour en sécuriser les sites stratégiques. Il est indispensable que les parties extérieures impliquées temporairement dans cette situation contribuent à la désescalade des tensions puis se retirent, dans le respect du calendrier indiqué publiquement par les autorités du Kazakhstan. Jean-Yves Le Drian s'est entretenu de cette crise avec Josep Borrell et, en tant que titulaire de la présidence du Conseil de l'Union européenne, la France maintiendra un dialogue étroit avec le Service européen pour l'action extérieure ainsi qu'avec ses partenaires de l'Union. Le Kazakhstan est un partenaire important de l'Union et de la France- vous avez rappelé mon déplacement en mai dernier dans

Madame la ministre, la violence se banalise dans notre pays : parmi les victimes de cette violence en constante augmentation figurent les maires et les élus. Entre janvier et novembre derniers, 1 186 élus, dont 162 parlementaires et 605 maires et adjoints, ont été victimes d'agressions physiques. Chacun, dans cet hémicycle, Chacun, dans cet hémicycle, connaît dans son département des élus qui ont été insultés ou menacés. Plusieurs élus reçoivent régulièrement des lettres de menaces destinées à les intimider. Le président Larcher a souhaité que le Sénat se constitue systématiquement partie civile lorsque

sans grand effet, car les poursuites ne sont pas systématiques et bien peu d'élus agressés sont informés des suites réservées aux affaires qui les concernent. Madame la ministre, quelles mesures concrètes comptez-vous prendre pour faire diminuer le nombre d'agressions et faire en sorte que les statistiques évoluent enfin dans le bon sens

en début de semaine, M. le Président de la République s'est lui-même exprimé sur le sujet pour faire part de son indignation et de son soutien à l'ensemble des élus qui ont vécu ces agressions, comme nous l'avions fait nous-mêmes.

qui a réaffirmé avec tous les présidents de groupe constitué qu'aucun débat démocratique ne pouvait se dérouler sous la menace. M. le président Gérard Larcher ici présent et vous tous partagez pleinement cette volonté d'apaisement du débat public,

Or, malheureusement, ce résultat est aujourd'hui inexistant. La parole est à M. Patrice Joly, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Monsieur le ministre, l'effondrement de la biodiversité et le réchauffement climatique deviennent des sources majeures d'instabilité, dans un contexte de montée des inégalités et d'effritement de la cohésion sociale. Il devient, en conséquence, impératif d'accélérer les transitions. L'objectif a été clairement défini : il nous faut baisser d'ici à 2030 nos émissions de gaz à effet de serre de 55 % par rapport à 1990. Cela ne se fera pas par magie. Il est demandé des efforts d'investissements massifs aux entreprises qu'aux ménages, en vue de décarboner le mode de vie de notre société et de réduire notre dépendance aux énergies fossiles, au moment où l'inflation pèse lourdement sur le pouvoir d'achat des ménages et asphyxie nombre de nos entreprises. Monsieur le ministre, le remboursement des emprunts réalisés pour financer les plans de relance et les dizaines, ou plutôt les centaines, de milliards d'euros d'investissements indispensables pour relever les défis climatiques et numériques en mettant en oeuvre des transitions socialement justes et soutenables requièrent des moyens importants, qui ne seront pas couverts par les nouvelles ressources propres de l'Union européenne. En effet, ces trois nouvelles ressources ne devraient produire en moyenne que 17 milliards d'euros par an d'ici à 2030 ; on est donc loin du compte ... Cela doit conduire à revenir sur les règles budgétaires européennes. Je pense aux référentiels relatifs à l'endettement- les fameux 3 % et 60 % du PIB issus du pacte de stabilité et de croissance

son propos à ce sujet a paru très évasif des comptes publics. Monsieur le sénateur Joly, vous m'interrogez sur le cadre budgétaire européen : sur les règles qui régissent son fonctionnement mais également sur les nouvelles ressources dont l'Union a décidé de se doter. de se doter. Je répondrai en trois points. En premier lieu, le simple fait que l'Union européenne ait décidé, il y a un peu plus d'un an, de se doter de nouvelles ressources propres, à la fois pour financer le remboursement des emprunts contractés solidairement

pendant l'année 2022, priorité étant donnée au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, au système d'échange de quotas. En deuxième lieu, nous savons qu'il faut « croiser », si vous me permettez cette expression, le débat sur la fiscalité internationale et les minima de taxation avec l'accord intervenu au sein de l'OCDE (Organisation de coopération et de dire que cet accord conclu au sein de l'OCDE sur une fiscalité minimale est la démonstration que les combats les plus longs peuvent être gagnés ; personne n'aurait imaginé, voilà quelques mois ou quelques années, que nous puissions collectivement aboutir à un tel accord sur la fiscalité minimale imposée aux multinationales.

et a posé quelques principes pour encadrer le débat qui va se dérouler tout au long du premier semestre de 2022. Le premier principe est celui de la crédibilité ; il faut que les règles qui encadrent l'évolution des finances publiques en Europe garantissent la crédibilité de notre économie et de notre monnaie.

de ces règles que la reconstruction européenne a pu être menée à bon rythme après la Seconde Guerre mondiale. Or c'est la perspective d'un investissement d'une ampleur analogue qui se présente à nous.

pour 2022 ... Il a tout de même trouvé le temps de déclarer dans la presse, en début de semaine : « Nous ne pouvons pas garder une balance commerciale déficitaire, car [ ...] c'est le reflet de la faiblesse de notre économie intérieure.

grâce à l'engagement et à la résilience des chefs d'entreprise, qui ont l'esprit de conquête, sont tournés vers l'international et ont, malgré les difficultés du fret maritime et de la crise covid,

qui procède de la consommation issue, en partie, de l'extérieur de notre pays et qui crée des besoins pour notre industrie en matière de composants, ce qui augmente mécaniquement

des matières énergétiques, en particulier du pétrole. Ainsi, la différence entre la hausse des exportations, dans un certain nombre de secteurs importants, et l'augmentation plus importante des importations creuse le déficit commercial des biens. C'est un élément conjoncturel. D'un point de vue structurel, le Gouvernement est à la tâche pour réduire ce déficit au travers de l'amélioration de la compétitivité du pays, de sa réindustrialisation, d'une politique commerciale

un nouveau protocole sanitaire à l'école a été annoncé ; c'est le troisième en moins d'une semaine. Il y a un an, personne n'était vacciné et les enfants n'étaient pas testés ; aujourd'hui, tout le monde est vacciné, les enfants sont testés. Les classes ont été fermées pour un cas positif, puis pour trois cas et maintenant on ne les ferme plus. On isolait les familles ; c'est fini. Les autotests n'étaient pas fiables ; ils le sont devenus.

de l'incertitude d'être accueilli à l'école. Vous avez annoncé un nouveau protocole, mais il n'est toujours pas publié ! Aussi, monsieur le ministre, quand cesserons-nous de naviguer à vue, avec des protocoles inadaptés ?

Nous aimerions tous que ces inconvénients n'existent pas, mais, s'il est assez facile de les décrire, il est évidemment plus difficile de les gérer et de « piloter à vue ». Je reprends votre expression, oui, en effet, le virus oblige la France, comme d'autres pays, à piloter à vue, c'est-à-dire à regarder ce qui se passe concrètement et à définir une réponse adaptée. Les évolutions que vous avez décrites

évidemment, c'est difficile. Bien sûr, il y a des souffrances au quotidien. Bien entendu, les tests nasopharyngés pour les enfants ne nous plaisent pas ; ils ne plaisent pas plus à moi qu'à vous et j'aimerais bien que cela n'existe pas, mais nous nous référons aux autorités de santé, nous étudions ce qui se passe dans le monde et, croyez-moi, nous n'avons pas à rougir de notre bilan. Ce qui me frappe au contraire, c'est cette volonté de toujours relativiser ce bilan, alors qu'il est internationalement reconnu que la France est le pays ayant réussi cette politique de l'école ouverte, grâce à nous tous, collectivement, grâce au pays entier. Pourquoi ne sommes-nous pas capables, toutes travées confondues, de développer une fierté nationale autour de ce bilan et de continuer dans cette phase, qui sera, je l'espère, la dernière ?

En application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des lois a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable- 23 voix pour, 2 voix contre -à la nomination de M. Didier Leschi à la direction générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, conformément aux mêmes dispositions, la commission des affaires économiques a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable- 12 voix pour, 10 voix contre -à la nomination de M. Benoît Coeuré à la présidence de l'Autorité de la concurrence. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (projet n° 327, texte

pénétrer dans les lieux publics pour éviter tout risque de propagation du virus. Dès lors, on peut considérer que seuls les détenteurs d'un test virologique répondent à cette exigence, à l'inverse des personnes vaccinées, dont il est aujourd'hui prouvé qu'elles peuvent être à la fois contaminées et contaminantes.

des programmes de rappel sans discernement ont toutes les chances de prolonger la pandémie, plutôt que d'y mettre fin ». À cet égard, les annonces du ministre français de la santé, imposant une dose de rappel d'abord

Alors que les évaluations de sécurité et d'efficacité des fabricants n'ont pas été menées à leur terme en ce qui concerne la troisième dose, il est nécessaire d'empêcher que ce passe vaccinal puisse être conditionné à l'administration de quatre, cinq, voire plusieurs autres injections, espacées de seulement quelques mois, comme l'a laissé entendre récemment le ministre des solidarités et de la santé. Le vaccin contre la grippe, virus qui mute régulièrement, est limité à une injection par an. D'autres vaccins nécessitent des rappels espacés de dix ans. L'administration d'autant de doses, dans des intervalles aussi courts, à une grande majorité de la population, constituerait une première. Il ne serait pas raisonnable de soumettre les Français à un tel rythme vaccinal, qui plus est quand leur emploi et leur vie sociale,

peut déterminer à l'avance le nombre de doses nécessaires pour assurer le maintien d'une protection suffisante contre le covid.

à un horizon de six mois ou un an. J'espère vivement, compte tenu du comportement du variant omicron, que la question ne se posera pas.

à ceux qui tiennent ces propos. Depuis quelques jours, le directeur de l'institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée, le professeur Raoult, tient des propos qui discréditent le vaccin. cet institut est largement financé par des fonds publics. Il devrait être le vaisseau amiral des maladies infectieuses en France, or c'est la boussole qui indique le sud ! Le maintien

pas qu'il ne faut pas vacciner pour protéger les populations. C'est l'inverse ! Il faut vacciner pour protéger l'ensemble des populations, nos populations et celles des pays qui n'ont pas les moyens de se payer ces vaccins.

Vous avez dit, monsieur le rapporteur, que ces amendements avaient le mérite de poser un débat. Justement, je souhaiterais profiter de la présence du ministre de la santé pour avoir ce débat. Il s'agit de la définition du schéma vaccinal complet.

qui nous a permis d'éviter que des pans entiers de la population soient décimés, considérant la contagiosité des variants ayant succédé au premier covid-19 et l'agressivité, notamment, du variant delta. Je peux considérer sans grand risque de me tromper, puisque ce n'est pas le ministre de la santé français qui vous le dit, mais l'ensemble des ministres au niveau planétaire et, surtout, des scientifiques, que si nous n'avions pas eu ce vaccin, que certains regardent avec un peu de dépit ou de lassitude, nous aurions eu beaucoup plus

mettez-vous dans la situation de quelqu'un qui fait des infections urinaires à répétition. Première infection, il prend un antibiotique et guérit. Trois mois plus tard, deuxième cystite, il prend des antibiotiques et guérit.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

je fais, depuis, des sérologies tous les deux mois. Et mon taux d'anticorps reste curieusement, mais heureusement, très élevé. Il est même indiqué, dans les résultats que je reçois, que mon taux d'immunoglobuline G (IgG) « témoigne du caractère récent de l'infection par le SARS-CoV-2 ou du résultat d'une vaccination récente ». Pourtant, dans quelques jours, sept mois après ma vaccination, mon passe ne sera plus valide et je vais devoir me faire vacciner à nouveau si je veux qu'il soit réactivé. Monsieur le ministre, je vous l'avoue, je ne suis pas très motivée Les experts constatent tous que le surdosage a pour effet d'augmenter les risques d'effets indésirables liés à la vaccination. La non-prise en compte de cette possibilité, qui est reconnue en Suisse, à cinq kilomètres de chez moi, m'interpelle.

sens : appliquer le principe de précaution, comme le font nos voisins helvétiques, qui ne sont pas des novices en matière d'expertise pharmaceutique.

suffisamment précisément, et tous les savants qui sont parmi nous pourront ensuite le corroborer. En réalité, quand vous avez été malade, vous pouvez avoir des anticorps, mais ces anticorps ne disent rien

qui sont capables, lorsque vous êtes exposé au virus et lorsqu'il « entre », de fabriquer des armes pour le bastonner et l'empêcher de se multiplier, donc de provoquer une infection- d'où la prévention des formes graves. Si, à la suite d'une prise de sang, on constate que vous avez des anticorps, c'est que, vraisemblablement, ou vous avez été exposé au virus ou vous avez été vacciné, ou les deux.

L'immunité cellulaire, elle, on ne peut en juger par une prise de sang. Ce n'est pas un taux d'anticorps : la capacité de vos cellules à réagir en cas d'agression, on ne peut pas l'estimer. Or, comme je vous l'ai dit, c'est bien l'immunité cellulaire qui entre en jeu, en cas d'infection, pour éviter qu'elle ne s'aggrave.

Comme médecins, nous utilisons les taux d'anticorps pour savoir si un malade a été infecté ou non, tout simplement. Mais il s'agit d'une notion plus qualitative que quantitative : la quantité d'anticorps n'a en réalité aucune importance

Or je me pose des questions quand j'observe un pays comme la Suisse, où l'on ne trouve pas seulement de l'argent : tous les laboratoires ont leur siège social en Suisse. Mon sentiment est que les lobbyistes de ces laboratoires ont influencé les parlementaires suisses qui ont décidé d'instaurer un passe sérologique.

: La parole est à Mme Sylviane Noël. Dans sa grande sagesse, le législateur avait prévu, à l'article 1 de la loi du 31 mai 2021, de sanctionner d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait d'exiger d'une personne la présentation d'un résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 en dehors des cas prévus par la loi. Dans une démocratie, la liberté est la règle, la restriction l'exception. Or il est particulièrement surprenant, et même inquiétant de constater que le présent texte prévoit la suppression de cette sanction.

notre assemblée s'était honorée d'adopter une disposition similaire, sur l'initiative de notre collègue Savin, exemptant de passe sanitaire la pratique d'une activité sportive. C'est un peu le même principe

l'exigence du passe vaccinal serait à géométrie variable. Comme si l'intérêt de la compétition l'emportait sur l'intérêt de l'exemplarité, auprès des jeunes et moins jeunes générations, du comportement que l'on peut attendre d'un grand sportif. Quelles sont en effet les valeurs du sport, sinon celles du dépassement de soi-même, de l'effort, de la fraternité ? Tous ces éléments me paraissent militer en faveur du maintien de la règle, et peut-être plus encore pour eux que pour les autres. C'est pourquoi, mon cher collègue- pardon d'y mettre de la flamme, mais je crois que le débat mérite d'avoir lieu -, je préférerais

il apparaît nécessaire et indispensable de rappeler le principe de l'égalité devant l'accès aux soins pour toutes et tous, sans discrimination. D'ailleurs, pour le docteur Patrick Bouet, médecin généraliste et président du Conseil national de l'Ordre des médecins, de la République ont permis à certains de laisser entendre qu'« un habitant de notre pays, parce qu'il a fait le choix de ne pas se faire vacciner, devrait alors se contenter de soins dégradés, faisant fi de son humanité intrinsèque pour n'être plus considéré

considéré qu'une stratégie de vaccination basée sur les rappels des premiers vaccins avait peu de chances d'être appropriée ou viable.

Monsieur Savary,

les exploitants qui ne contrôleraient pas correctement le passe vaccinal de leurs clients. Cet amendement propose de supprimer cette disposition qui est disproportionnée. En effet, la loi fait déjà peser sur les exploitants la lourde responsabilité de contrôler les données de santé de leurs clients. Depuis le début de la crise sanitaire, les restaurateurs ont joué le jeu ; ils ont lourdement payé les conséquences de cette crise par de longues périodes de fermeture et l'imposition de jauges. Personnellement, je regrette que ce texte soit si répressif. Aucun exploitant n'a intérêt à avoir un cluster dans son établissement. Il faudrait pouvoir laisser davantage de place à la confiance.

l'obligation pour les établissements de contrôler leurs clients transforme substantiellement leur quotidien. Il est contre-productif d'accabler des professionnels déjà acculés par la crise sanitaire et de faire preuve de défiance à leur égard, d'autant plus que la plupart d'entre eux jouent le jeu avec beaucoup de résilience depuis le début de la pandémie. En tout état de cause, ces nouvelles sanctions contreviennent au principe de proportionnalité des peines, qui soumet le droit pénal français au principe selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires.

Outre le caractère complètement disproportionné de l'amende de 10 000 euros qui est prévue, il n'est pas acceptable que les professionnels, déjà largement touchés par la crise depuis maintenant près de deux années, soient victimes de la politique sanitaire défaillante du Gouvernement. Pour rappel, ces professionnels ont connu des fermetures, des jauges, des couvre-feux, sans compter les investissements qu'ils ont dû réaliser pour se mettre aux normes et protéger leurs clients. Dans la société du contrôle de tous par tous que le Gouvernement souhaite instaurer, il n'est pas admissible que les professionnels, sur lesquels l'État se décharge pour opérer ses missions de contrôle, doivent subir des sanctions aussi importantes. Nous demandons donc le maintien des sanctions

Le projet de loi sanctionne tout manquement du responsable de l'établissement constaté à plus de trois reprises dans un délai de trente jours à six mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende. Ces sanctions sont définies par référence à celles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique. Ce renvoi au quatrième alinéa est supprimé par l'amendement. Le renforcement des sanctions est déjà assuré par le projet de loi, dès lors qu'il est envisagé une amende prévue pour une contravention de la cinquième classe dès le premier manquement.

En outre, la sanction la plus dure dans cette situation repose sur la décision de fermeture administrative de l'établissement- une sanction extrêmement lourde. Par conséquent, le cumul du risque de fermeture de l'établissement et d'une amende de cinquième classe dès la première infraction constatée s'avère strictement nécessaire, proportionné et adapté aux risques sanitaires encourus sans qu'il soit utile d'en rajouter.

des sanctions susceptibles d'être infligées à un responsable d'établissement, dont l'accès est assujetti à la présentation du passe sanitaire, qui n'aurait pas rempli ses obligations légales de vérifier que les personnes qui accèdent à son établissement

une mise en demeure et, si le chef d'établissement ne s'y conforme pas immédiatement, la sanction est la fermeture temporaire de l'établissement.

il nous semble qu'inciter les gens qui souhaitent se faire vacciner, même après avoir fait un choix contraire, est une bonne chose. Le dispositif du repentir permet de répondre aux situations dans lesquelles une personne est désormais prête à se faire vacciner, mais n'ose pas se manifester de peur des sanctions qu'elle encourt.

déclinaison d'une politique pénale mise en oeuvre avec les parquets et la seconde consistait à fixer clairement une règle juridique d'extinction de la peine.

qui, j'y insiste, n'est pas obligatoire, et il a des sanctions pénales. Pourtant, ils ont commis l'un et l'autre la même faute. Telle n'est pas la conception que j'ai du droit pénal et telle n'est pas la conception que la commission des lois a du droit pénal. L'avis est donc très fermement défavorable.

par l'Assemblée nationale, sur la proposition de M. Guillaume Larrivé, et qui prévoyait la possibilité pour les organisateurs de réunions de campagne de l'élection présidentielle non seulement d'en restreindre l'accès

il ne fallait pas non plus que ce soit un barrage à l'accès de nos concitoyens à ces événements. Il importe quand même que la liberté d'opinion puisse se manifester

En effet, il n'y a pas lieu de différencier le régime de l'accord parental suivant que le mineur concerné par la vaccination contre le covid-19 a entre 5 et 11 ans ou entre 12 et 16 ans.

Alors que la vaccination est désormais ouverte à l'ensemble des enfants âgés de 5 à 11 ans, celle-ci est subordonnée à la présence d'au moins un parent accompagnateur, ainsi qu'à la remise au personnel du lieu de vaccination d'un formulaire d'autorisation parentale rempli et signé par les deux parents. Or, chacun peut l'imaginer, le fait d'exiger l'accord des deux parents peut être une source de difficultés importantes au sein des familles, cristallisant potentiellement des désaccords et des conflits profonds entre les parents, alors qu'il y a lieu de dédramatiser cet événement et de rendre la vaccination plus rapide et plus facilement accessible. En plus de ces considérations, qui relèvent de l'intimité des familles, il faut avoir à l'esprit les difficultés pratiques et judiciaires que pourrait que pourrait susciter cette obligation, avec notamment un risque d'engorgement du côté des juges aux affaires familiales. Nous avons déjà été alertés sur ce point. L'objet de cet amendement est donc de réduire les contraintes concernant la vaccination des mineurs de 5 à 11 ans en l'alignant sur le régime des mineurs âgés d'au moins 12 ans, à savoir

très clair : entre 16 et 18 ans, le mineur a le droit de se faire vacciner sans avoir à demander la permission de ses parents ; entre 12 et 16 ans, il peut être vacciné dès lors qu'un des deux parents

ce principe, on finit par créer de grandes difficultés. Si on le fait pour le vaccin, qui n'est pas indispensable pour les tout-petits, alors,

Merci En juillet dernier, lors des débats sur la précédente loi de gestion de la crise sanitaire, j'avais plaidé pour l'adaptation des mesures au contexte sanitaire et social des territoires d'outre-mer. Je n'avais pas été suivi, monsieur le rapporteur. Je me félicite de voir qu'aujourd'hui le texte adopté par l'Assemblée nationale et modifié par notre commission des lois prévoit cette possibilité d'adaptation locale. Fort heureusement, dirais-je, car la population de la Guyane et des Antilles est deux fois moins vaccinée que la population de l'Hexagone. Pour des raisons culturelles et historiques, les décisions touchant aux libertés publiques y sont accueillies avec beaucoup de méfiance, pour ne pas Il en a résulté une application difficile du passe sanitaire, et il a fallu de la pédagogie aux autorités locales pour commencer à le voir accepté. Au quotidien, il suscite cependant encore beaucoup d'oppositions. C'est pourquoi il me semble compliqué, voire impossible, d'appliquer le passe vaccinal dans les mêmes conditions que dans l'Hexagone. Les tensions sont encore très vives et nous devons éviter de pousser une frange de la population vers l'insurrection. Nous sommes dans un entre-deux. Compte tenu de l'ampleur des contaminations, la seule mesure efficace pour venir à bout de cette épidémie et du variant omicron serait un confinement strict. Certes, la vaccination est l'outil le plus efficace actuellement à notre disposition, mais, en attendant une amélioration des taux de couverture vaccinale, je propose d'aller un peu plus loin que le texte de la commission dans les possibilités d'adaptation offertes aux représentants de l'État dans les régions et départements d'outre-mer. Ainsi, je souhaite que soit maintenu le passe sanitaire, partiellement ou totalement, en lieu et place du passe vaccinal, sans autre limite que sa durée d'application. Cela offrira toute la souplesse nécessaire pour s'adapter aux situations locales, notamment celles, particulières, des Antilles et de la Guyane.

l'instruction de différer l'entrée en vigueur de la loi. J'ai considéré que, sur le plan de la mécanique, c'était tout à fait impossible. En effet, quand la loi est votée par le Parlement, elle s'impose à tous.

serait une incongruité constitutionnelle : la Constitution est tout de même là pour faire en sorte que la loi soit la même pour tous Pour autant, j'ai bien compris ce qui motive chacun de ces amendements, à savoir la situation particulière de nos collectivités d'outre-mer. Nous avons déjà rencontré ce problème tout

d'entrée en vigueur de la loi, qui, elle, relève de l'application de principes constitutionnels. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer vos amendements, si j'ai réussi à vous persuader. À défaut, je serai obligé de donner, au nom de la commission, un avis défavorable.

Je ne peux qu'émettre un avis favorable sur cette proposition. La rédaction qui a été retenue par la commission est plus contraignante en ce qu'elle limite, d'une part, le pouvoir d'adaptation du préfet uniquement au passe sanitaire, et, d'autre part, la durée pendant laquelle le représentant de l'État peut adapter les mesures. La situation propre à chaque territoire ultramarin nécessite que les représentants de l'État disposent d'une palette d'actions suffisamment large pour pouvoir faire face à chaque situation et elle implique que les préfets puissent adapter régulièrement les mesures prises afin d'aboutir progressivement à la mise en place de ce passe vaccinal sur tous les territoires. Il est évident que nous visons le même but, peut-être avec une

c'est que la gestion d'une telle crise sanitaire dans les territoires ultramarins nécessiterait une différenciation que ne permettent pas les statuts actuels de ces territoires.

ont eu une autre approche de la gestion de l'épidémie. La Nouvelle-Calédonie a ainsi appliqué du « zéro covid » jusqu'au mois d'août dernier, lorsqu'un jugement

compliquées. La nouvelle direction générale du CHU de Martinique, l'ARS et le préfet ont mis en place des instances de conciliation, qui sont en train de faire un travail pour amener petit à petit, mais le plus rapidement possible, les soignants

en refusant celle que je vous ai proposée et dont je suis certain à la fois qu'elle aura le même effet utile et qu'elle est constitutionnelle, alors vous prendrez un risque. Si vous considérez que cela vaut le coup, prenez-le

Par un parallélisme des formes qui ne surprendra personne ici, nous demandons dans cet amendement la suppression de l'état d'urgence sanitaire à la Réunion et à la Martinique, suivant la logique qui nous a conduits,

l'état d'urgence sanitaire avant le 1 mars 2022 dans une autre collectivité ultramarine que celles dans lesquelles il est prorogé par le présent projet de loi, cet état d'urgence serait également prorogé jusqu'au 31 mars

? Il est défavorable sur ces deux amendements. Je crois que le Gouvernement fait bien de maintenir l'état d'urgence sanitaire dans un certain nombre de collectivités où l'épidémie suscite de très graves inquiétudes. En revanche, madame la ministre, c'est délibérément que nous n'avons pas voulu vous permettre de déroger à la loi

à cette date, puisque c'est plutôt dans les collectivités où l'état d'urgence sanitaire s'exerce déjà qu'on a de bonnes raisons de penser qu'il pourrait être nécessaire de le proroger. Dès lors, pourquoi voulez-vous inscrire

L'hôpital fait aussi et surtout face à un important manque de moyens humains. Ce manque de personnel met en danger les soins assurés à nos concitoyens ; il met aussi à l'épreuve les soignants restants, qui doivent assumer l'obligation de soins avec moins de moyens.

sont fatigués. » Ces héros, ce sont nos soignants ! J'ai expliqué tout à l'heure pourquoi il valait mieux quelqu'un de vacciné positif plutôt qu'un non-vacciné avec un test négatif à un instant t ; je ne recommencerai pas cette explication. Pour nos héros, pour nos soignants, maintenons la vaccination : il faut être vacciné, et non pas

Par cet amendement, nous souhaitons subordonner l'entrée en application du nouveau passe vaccinal à la démonstration de l'efficacité du passe sanitaire.

« sur la nécessité que les éléments qui permettent d'apprécier l'efficacité des traitements susmentionnés lui soient rapidement transmis, afin de continuer l'exercice de sa mission

publication de cet avis. À cet égard, elle rappelle que « l'utilisation des dispositifs précités reste conditionnée à des garanties relatives à leur efficacité

En un an, les chiffres parlent d'eux-mêmes : 74 % de tous les vaccins fournis l'année dernière sont allés vers des pays à haut revenu ou de la tranche supérieure Moins de 1 % d'entre eux sont allés vers des pays à bas revenus. Je veux faire un petit rappel : en France, 87 % de la population est vaccinée ; au Nigéria, ce taux est de moins de 2 % ! Je sais que le Gouvernement oppose à la levée des brevets le mécanisme Covax. De fait, ces deux systèmes ne s'opposent pas, mais il convient de reconnaître que la France se trouve dans le haut du classement parmi les pays donateurs, en compagnie notamment des États-Unis, de la Chine et du Japon. En effet, le Gouvernement indique que 67 millions de doses

de ces initiatives : au rythme actuel, ce n'est qu'en août 2024 qu'un taux de vaccination de 70 % sera atteint ; cela reste insuffisant. La santé est un droit qui doit être assuré par des mesures politiques ; la levée des brevets avec

En effet, les débats parlementaires ont pris du retard. Il nous semble donc nécessaire de décaler l'instauration de ce passe vaccinal. Si l'on tient compte des délais d'obtention des rendez-vous

Il nous semble donc absolument nécessaire, y compris par rapport au contenu plutôt liberticide de ce passe vaccinal, de laisser aux personnes qui le souhaitent le temps de se faire vacciner. la mise en place de ce dispositif doit aussi,, être accompagnée d'un renforcement de la campagne vaccinale, ce qui s'avérera impossible

servir du présent texte pour donner au Gouvernement des moyens de convaincre nos partenaires européens de prendre des décisions qui vont s'appliquer à des entreprises américaines, sur les brevets de vaccins. Je comprends bien votre intention, que je partage d'ailleurs

à accepter, d'autant que je ne vois pas quel effet aurait sur nos partenaires la menace de ne pas appliquer le passe vaccinal en France s'ils ne nous cédaient pas sur l'accès des pays pauvres à la vaccination. L'avis de

au service de toutes les populations, sans discrimination sociale ou territoriale, à l'échelle de la planète. Enfin, bien évidemment, se pose la question de la maîtrise des données et du contrôle d'un certain nombre de règles de droit. Certes, ce ne sont pas

Tedros Adhanom Ghebreyesus, nous déclarait dès le mois de mai : « Il n'y a pas de manière diplomatique de le dire : un petit groupe de pays qui fabriquent et achètent la majorité des vaccins contrôlent le sort du reste du monde. »

à avancer dans cette discussion pour aboutir à la levée des brevets sur les vaccins. Cela doit être l'un des objectifs prioritaires d'Emmanuel Macron, qui nous a lui-même affirmé qu'il était tout à fait favorable à ce que la propriété industrielle soit levée sur les vaccins contre Oui, nous devons faire de ce vaccin un bien public, un bien commun mondial

restant en discussion des propositions de loi ordinaire et organique relatives aux lois de financement de la sécurité sociale ne sont pas parvenues à l'adoption d'un texte commun.

J'informe le Sénat que deux candidatures, en remplacement de deux membres démissionnaires, pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire